illégale passe par des installations ne respectant pas, bien entendu, les normes sociales et environnementales, ce qui permet de proposer aux détenteurs de ces véhicules des prix d'achat plus attractifs.

ce qui porte atteinte à l'environnement et aux emplois de cette filière. Pour autant, la mesure que vous proposez me semble porter sur un périmètre trop large, ce qui alourdirait par trop la charge administrative des assurances et des automobilistes. En effet, cinq millions de contrats d'assurance automobile sont résiliés chaque année

détruit. Il serait utile de mieux cibler la mesure, comme y tend l'amendement n° 597, qui vise la situation des véhicules accidentés irréparables, soit 200 000 cas de résiliation par an, dont près de la moitié des propriétaires refusent de céder le véhicule à l'assurance.

Cette filière vise à offrir aux particuliers et aux collectivités la possibilité de procéder au traitement des bateaux hors d'usage qu'ils détiennent.

étaient distribués gratuitement le long des routes aux enfants. Depuis lors, la consommation de chewing-gums, de la gomme à mâcher, a explosé dans le monde. En effet, près de 100 kilos de chewing-gums sont consommés chaque seconde, pour quelques minutes de dégustation. Ces Ces chewing-gums constituent une source de pollution : ils ne sont biodégradables qu'au bout de cinq ans et se retrouvent souvent jetés dans la nature, désagrégés en microparticules. représentent un coût élevé pour les collectivités territoriales, une perte d'énergie et de temps, puisqu'il faut utiliser des jets d'eau chaude à très haute pression pour les retirer des trottoirs, des rues ou autres couloirs de métro. Il s'agit du deuxième déchet le plus produit au monde après les mégots de cigarette, qui feront l'objet d'une filière REP à compter du 1 janvier 2021. Les chewing-gums, semble-t-il, peuvent peuvent être valorisés pour fabriquer des semelles de chaussure. Les producteurs pourraient dès lors contribuer à leur collecte et à leur recyclage via leur contribution. Dans tous les cas, il est préférable de les intégrer à la conception de chaussures plutôt que de les retrouver englués à nos semelles ou sur les trottoirs ! Le présent amendement vise essentiellement à appliquer le principe du pollueur-payeur en créant une filière REP pour les gommes à mâcher synthétiques.

parole est à M. Frédéric Marchand. Nous avons fait partie de ceux qui, en commission, ont permis, par la voie de leur amendement, d'étendre la filière REP lingettes à l'ensemble des textiles sanitaires. L'extension du périmètre de la REP des lingettes pré-imbibées pour usage corporel et domestique aux textiles sanitaires n'a pas encore donné lieu à une étude d'impact. Or elle pourrait conduire à une hausse du prix des produits de première nécessité, dont les couches, qui représentent un budget significatif pour les familles les plus modestes. Une réflexion devra être menée avant les débats à l'Assemblée nationale sur la mise en place, dans le cadre du principe du pollueur-payeur, d'un système de collecte et de traitement des déchets issus de certains textiles sanitaires utilisés dans des établissements où une massification des flux semble possible. Cette réflexion devra prendre en considération les impacts en termes de développement industriel d'une telle filière. Quel est l'avis de la commission La commission a étendu la filière REP lingettes à l'ensemble des textiles sanitaires. Et pour cause ! Les textiles sanitaires représentent un gisement de déchets non recyclables considérable et un poids pour les collectivités et, donc, pour le contribuable. L'intégration de ces textiles à une filière REP doit permettre d'améliorer l'éco-conception et d'orienter les producteurs vers des solutions alternatives. que ces produits représentent un budget important pour les familles. Cependant, ce texte de loi ne doit pas perdre de vue son ambition environnementale. Les questions sociales doivent être traitées dans un autre cadre que ce texte, même si, bien évidemment, et nous le partageons, cher collègue, ce sont des considérations très importantes pour nous

Nous le savons, elles constituent une source importante de déchets, car elles sont impossibles à recycler et sont donc traitées avec les ordures ménagères résiduelles. représentent un coût important pour les collectivités chargées du traitement de l'eau, puisqu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts aux canalisations. Cet amendement vise donc à avancer de trois ans la date d'application du principe pollueur-payeur aux textiles sanitaires, y compris aux lingettes pré-imbibées.

Mme la rapporteure. Une entrée en vigueur en 2021, ainsi que vous le demandez, de cette nouvelle REP semble trop anticipée.

Le polystyrène est l'un des matériaux les moins recyclés et recyclables sur le marché. Actuellement, cette résine plastique focalise l'attention et les critiques dans le cadre de l'extension des consignes de tri à tous les emballages : elle est difficile à séparer des autres résines utilisées pour les emballages ; il n'existe pas de filière de recyclage en France ; elle représente des volumes importants. se retrouve partout dans de nombreux produits quotidiens, tels que les pots de yaourt. Cela peut sembler anodin, mais on jette en France seize milliards de pots de yaourt par an, alors même qu'on ne sait pas les recycler, car ils sont majoritairement faits de polystyrène. Ainsi, l'industrie des produits laitiers représente 40 % du montant du polystyrène. Ces pots de yaourt finissent enfouis ou incinérés, ce qui est un véritable désastre environnemental. Des réflexions sont en cours, notamment au sein du Syndicat national des fabricants de produits laitiers frais ou encore chez Saint-Gobain, pour créer une filière de recyclage sous l'impulsion de la feuille de route pour l'économie circulaire. Par cet amendement, nous vous proposons d'encourager ces premiers balbutiements

Cher collègue, aucune filière REP ne porte sur un matériau en particulier : les filières portent sur des catégories de produits. Je le regrette, mais cela est le fruit de la construction historique des filières REP. Il ne me semble pas opportun de remettre cet équilibre en cause. L'avis est évidemment défavorable. Quel est

Préville. Nous ne l'avons pas voulu, mais c'est un fait, une vérité crue et nue : si nous ne faisons rien, il y aura bientôt plus de plastiques dans les océans et les mers que de poissons.

Tout plastique rejeté dans la nature finit par y aboutir. Nous n'avons pas encore fini de découvrir l'étendue de ce désastre écologique, la quantité croissante de macroplastiques, de microplastiques Dernière découverte en date : la « plasticroûte » sur les roches de l'île de Madère. À peine avons-nous intégré les faits que d'autres s'ajoutent, encore plus graves à bien des égards. Cela s'apparente à une descente aux enfers. Nous nous devons d'agir et, point par point, de trouver des solutions multiples et variées qu'il faudra déployer pour remédier à cette pollution dans les mers et les océans. Chaque année, 800 tonnes de filets et 400 tonnes de chaluts usagés sont jetées, perdues ou abandonnées. Ils représentent une véritable pollution en mer et figurent en troisième position du top dix des déchets de ressac. Les équipements de pêche représentent 70 % des déchets plastiques qui flottent à la surface des mers et des océans. Ils sont responsables de dégâts sur les habitats, les paysages sous-marins, mais, surtout, ces filets, qui mettent des années à se dégrader, sont responsables de la pêche fantôme, c'est-à-dire qu'ils continuent à piéger poissons et animaux marins pour rien. Ils peuvent être aussi ingérés par les mammifères marins : n'a-t-on pas retrouvé dans l'estomac d'un cachalot échoué plus de quinze kilogrammes de plastique, dont un filet de pêche de treize mètres de long ? Ainsi,

Si la directive sur les plastiques à usage unique prévoit bien une couverture des filets de pêche, les producteurs envisagent, pour l'heure, de mettre en place un système volontaire et non pas une REP, selon les informations que nous a transmises le Gouvernement. La transposition de la directive ne nécessiterait donc pas, à mon sens, l'inscription d'une REP supplémentaire à la liste prévue par la loi. Mais, pour en être parfaitement certains, nous allons demander l'avis du Gouvernement. Quel est La directive sur les plastiques à usage unique prévoit la mise en place d'une filière de collecte et de recyclage pour les engins de pêche et les équipements d'aquaculture d'ici à 2025. Pour ces produits uniquement, la directive prévoit que cet objectif puisse être atteint par la mise en place d'accords volontaires plutôt que par la création

Les objets de décoration, par exemple les décorations de Noël, sont souvent fabriqués à partir d'une multitude de matériaux assemblés : bois, plastique, paillettes, métal, etc. C'est un gâchis lorsqu'ils sont jetés gâchis de matériaux, produits toxiques, surcharge des poubelles grises ou noires, selon les cas, inutilement encombrées, d'autant plus que leur prix peu élevé dans un contexte de consommation effrénée est un véritable problème. Le coût écologique n'est pas marginal. La nocivité pour la santé et l'environnement est l'un des six critères retenus par l'Ademe pour justifier la création d'une REP. À titre d'exemple, les paillettes utilisées en décoration sont composées de plastique et d'aluminium liés à du polyéthylène

Avis défavorable. De nombreux produits de décoration sont des textiles ou des meubles qui relèvent déjà d'une filière REP existante. Créer une telle filière pour les autres articles de décoration, par exemple des bibelots ou des décorations

D'après le baromètre numérique 2018, 94 % des Français sont équipés d'un téléphone portable et 75 % plus spécifiquement d'un smartphone. Or le smartphone est par définition un produit dont le renouvellement est fréquent, conséquence d'une obsolescence programmée très répandue, mais aussi de la volonté des consommateurs de disposer des dernières fonctionnalités techniques. Plusieurs études, notamment de l'Ademe, ont mis en évidence le caractère polluant de ces produits, que ce soit en termes d'extraction des matières premières, de fabrication des composants ou de transport. Par ailleurs, des tonnes de smartphones usagés sont parfois acheminées illégalement vers des décharges situées en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est. Selon un rapport du programme des Nations unies pour l'environnement, plus de la moitié- entre 60 et 90 % -des déchets électroniques provenant d'Europe et d'Amérique du Nord échappent aux filières de traitement et sont enfouis ou vendus en Afrique, en toute illégalité. Pour Pour une question d'exemplarité et de responsabilité environnementale, la France doit absolument se saisir du sujet. Alors que la filière REP D3E englobe normalement ces déchets, seuls 15 % d'entre eux sont effectivement recyclés. C'est pourquoi je propose la création d'une filière REP spécifique aux téléphones mobiles et aux smartphones. Quel est l'avis de la commission ? Les téléphones mobiles et les smartphones sont aujourd'hui couverts par la REP D3E, vous l'avez rappelé. Il semble plus pertinent d'améliorer la collecte et la valorisation des téléphones dans ce cadre

dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant. Ces recettes financeraient la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et le développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d'inciter les metteurs sur le marché de ces produits à développer un peu plus l'éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l'atteinte de l'objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.

dont les recettes, collectées par un organisme indépendant, financeraient la création de nouvelles filières de collecte séparée de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. La commission est très réservée sur la pertinence d'un tel mécanisme. Premièrement, faute de filières REP spécifiques à ces produits, ces éco-contributions ne permettraient pas de financer directement l'amélioration de la prévention et de la gestion des déchets qui en sont issus. Elles viendraient simplement alimenter le budget de l'Ademe ou d'un autre organisme public. On aurait ainsi une éco-contribution commune sur des produits totalement différents, par exemple sur les livres ou sur des ballons de baudruche, qui ne sont pas couverts aujourd'hui par une filière REP. filière REP. Par conséquent, il serait très difficile de calculer cette éco-contribution commune sur une quantité de produits très divers. Deuxièmement, la mise en place d'une éco-contribution généralisée s'apparenterait en réalité à une taxation environnementale, puisqu'elle viserait indifféremment et uniformément des catégories de produits très diverses. La commission ne peut être que très réservée sur l'introduction d'une telle taxation environnementale, qui pèserait directement sur le pouvoir d'achat des Français. Troisièmement, en tout état de cause, si une telle option devait être envisagée, il serait préférable de prévoir la création d'une TGAP sur l'ensemble de ces produits

est à Mme Laure Darcos. Le principe de la responsabilité élargie du producteur vise à obliger les metteurs sur le marché à prendre en charge la gestion de leurs produits en fin de vie. Toutefois, ceux-ci ne peuvent pas être tenus pour responsables des dommages à l'environnement découlant des incivilités et des pratiques illégales auxquelles se livrent les utilisateurs de leurs produits.

En outre, alors même que les pouvoirs publics et les professionnels se battent au quotidien contre les trafics et les pratiques illégales qui touchent économiquement les filières et, bien sûr, portent cette disposition risque de décourager cette lutte : elle serait un blanc-seing pour les acteurs de pratiques illicites, puisque le financement de leurs dégradations et de leurs impacts sur l'environnement sera assuré par les professionnels respectueux de la légalité. Elle constitue donc un signal négatif profondément préjudiciable à l'ensemble des acteurs économiques en matière de préservation de l'environnement. Par ailleurs, cette disposition n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact, ni même d'une concertation avec les professionnels. Or, si elle était appliquée en l'état, elle pourrait engendrer des coûts majeurs pour les filières. amendement vise donc à exclure du principe de la REP le ramassage, le traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés et la dépollution des sols : il faut assurer un juste équilibre entre la responsabilité des metteurs sur le marché, celle des utilisateurs des produits et celle des personnes chargées de faire respecter la loi.

est de nature juridique : la directive sur les déchets ne permet pas d'ajouter une obligation qui pourrait ne pas être directement liée aux déchets issus de produits mis sur le marché par les contributeurs d'une REP.

à revenir sur cette modification. Les dépôts sauvages constituent un fardeau, non seulement environnemental, mais aussi financier pour nos territoires. Le coût de ramassage, de traitement des déchets, ainsi que de dépollution des sols est estimé, par une récente étude de l'Ademe, à plus de 300 millions d'euros pour les collectivités territoriales et leurs groupements ; on observe également de grandes différences entre les territoires. Il me semble indispensable que ces coûts, aujourd'hui supportés par les contribuables à hauteur de 5 euros par an et par habitant, soient pris en charge par les producteurs conformément au principe du pollueur-payeur, logique de la responsabilité élargie du producteur. Aussi, sur ces deux amendements, la commission se prononce défavorablement.

de produits en plastique, malheureusement trop souvent retrouvés dans l'environnement. Les collectivités territoriales supportent depuis trop longtemps les nuisances et les coûts de gestion de ces dépôts sauvages ; aussi, j'émets un avis défavorable

du traitement des déchets abandonnés ou déposés et de la dépollution des sols aux cas où il est établi que le metteur sur le marché n'a pas mis en oeuvre ses obligations propres à assurer une gestion adéquate de ses produits en fin de vie.

Mme Nicole Duranton. Les biodéchets représentent 30 % des déchets de nos poubelles et ne sont pas valorisés. Aussi, afin d'atteindre l'objectif de réduction des déchets tel que défini par le programme national de prévention des déchets 2014-2020, nous proposons d'encourager le tri des biodéchets et de les valoriser par méthanisation ou compostage. Il s'agit d'inciter les collectivités territoriales à développer des filières de compostage de biodéchets, y compris du tri sélectif, de la collecte, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage par l'octroi d'une incitation financière.

Les biodéchets, qui représentent un tiers des poubelles des Français, peuvent être utilement exploités pour enrichir les sols en matières organiques. Ils constituent une chance pour notre agriculture. Les plastiques biodégradables et compostables favorisent la collecte des biodéchets, car ils simplifient le geste de tri et facilitent le tri à la source. Ils sont orientés dans la même poubelle que les biodéchets et valorisés au même titre que ces derniers dans la filière de compostage. C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à réserver la part d'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de plastiques biodégradables aux collectivités qui souhaitent développer la collecte séparée des biodéchets pour un recyclage

ne contient pas de mesure spécifique relative à la gestion des biodéchets, tels que les déchets alimentaires, qui représentent 30 % à 40 % des poubelles résiduelles des ménages des Français. La loi de transition énergétique pour la croissance verte rend pourtant obligatoire le tri à la source des biodéchets avant 2025 ; ce tri est

soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets. Or, en droit français, aucune disposition ne permet à ce stade de préparer avec des moyens financiers cette future obligation. En conséquence, pour que le présent texte réponde pleinement aux objectifs de la feuille de route il est nécessaire d'encourager la mise en place de filières de recyclage des biodéchets par méthanisation ou par compostage, procédés permettant de produire de l'énergie et des amendements naturels de très haute qualité.

d'encourager la mise en place de filières de recyclage de biodéchets par méthanisation ou par compostage. En France, la recette de la collecte du « point vert », payée par les producteurs d'emballages, représente 800 millions d'euros environ. Cette somme est actuellement gérée par l'organisme Citeo. Les emballages plastiques biosourcés et compostables contribuent à hauteur de 1 % de cette collecte, ce qui représente environ 8 millions d'euros par an. Cette somme pourrait être réservée aux projets des collectivités qui souhaitent développer la collecte séparée des biodéchets

et 424 rectifié : cette proposition conduirait à segmenter les éco-contributions en fonction du mode de valorisation de chaque produit. Les éco-organismes sont des systèmes collectifs de gestion des déchets mis en place par les producteurs ; un tel découpage est concrètement irréalisable.

les contributions financières des producteurs doivent obligatoirement couvrir les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés, y compris lorsque ces déchets ont été abandonnés avant l'application à ces produits de la responsabilité élargie des producteurs. Ainsi, les metteurs Ainsi, les metteurs sur le marché de produits donnant fréquemment lieu à des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe du pollueur-payeur. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse planer un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être prise en charge.

totalement différent en fonction des territoires, nous proposons que chacun d'eux dispose d'une majoration propre prenant en compte ses particularités. En effet, un seul taux multiplicateur, prévu de manière un peu informe pour l'ensemble des collectivités d'outre-mer, ne saurait répondre à la situation de chaque territoire. Je Je vous demande tout simplement de donner du sens à la volonté de différenciation affichée en permanence par l'exécutif et, en particulier, par le Président de la République ! Karam. L'article 8 prévoit un dispositif de majoration des soutiens pour les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, dont les coûts observés sont supérieurs à ceux de l'Hexagone, compte tenu de l'éloignement et de l'insularité de ces territoires, ainsi que de la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont déployés. Je le disais il y a quelques instants : à mon sens, outre l'éloignement et l'insularité, l'enclavement de certains territoires ultramarins, en particulier la Guyane, doit être pris en compte dans ce dispositif de majoration. Les intercommunalités de l'est et de l'ouest guyanais, chargées de la gestion de sites particulièrement enclavés, cumulent les déficits structurels. Des évolutions du système de financement sont donc indispensables, notamment pour les zones les plus isolées et les plus précaires. Ces dernières n'ont pas la possibilité de transférer leurs déchets vers des centres de stockage autorisés à des coûts acceptables, ce qui entraîne la constitution de dépôts sauvages et un grave risque sanitaire. Pour cette raison, cet amendement vise à prendre en considération l'enclavement et les problématiques liées aux sites isolés dans le dispositif de majoration des soutiens à destination des collectivités territoriales ultramarines concernées.

ne disposent pas d'une compétence propre en matière d'environnement. Cependant, ces territoires sont confrontés aux mêmes problématiques que les collectivités de l'article 73 de la Constitution. Il convient donc d'étendre le champ d'application de cet article aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

le cadre juridique en vigueur prévoit déjà la consultation de la commission des filières REP et du Conseil national d'évaluation des normes. Les représentants des collectivités territoriales sont donc largement associés à ces travaux

adaptés aux emballages compostables. Il s'agit de faciliter le tri et de mettre fin à l'incinération ou à l'enfouissement de ces emballages faute de filière adaptée. de mélanger les emballages compostables et les biodéchets, on assurerait une économie de tri significative pour les collectivités et une simplification du geste pour le consommateur. Un pilote de test de collecte et de compostage industriel d'emballages en acide polylactique a été mis en place par Citeo à Paris à la fin de 2018. L'objectif est de certifier que le compostage industriel répond aux normes de qualité du compost et de trouver un mode de collecte adapté pour ces emballages.

Il ne nous semble pas opportun d'apporter une précision sur le sujet spécifique des emballages : on risquerait de complexifier davantage la mise en oeuvre de ce principe et de mettre en difficulté les principaux acteurs concernés. Aussi, la

Les producteurs de ces emballages n'ont pas encore créé une telle filière pour les déchets issus de leurs produits. Ces déchets ne sont donc pas valorisés actuellement. Cet amendement tend à imposer le déploiement par l'éco-organisme d'une telle filière, qui devra être financée par les producteurs de ces emballages.

de personnes sont conduites à faire. D'ailleurs, je prévois de saisir l'Anses des risques de dispersion de microplastiques dans l'environnement via le compostage de ces plastiques. Dans ce contexte, obliger au développement d'une filière de compostage industriel des emballages compostables ne me paraît pas opportun nous devons encore travailler sur l'impact de ces plastiques.

est la mise à contribution des acteurs du secteur, par le biais des sommes qu'ils versent d'ores et déjà aux éco-organismes.

d'État. Il ne me semble pas pertinent de définir, comme vous le proposez, un moyen financier déconnecté de tout objectif. Je suis totalement d'accord avec vous, le but, c'est de développer l'économie de la fonctionnalité, mais, de

une question d'usage qui fait partie de l'économie de la fonctionnalité. Autour de tels modèles doivent se développer des innovations inhérentes à ce type de nouvelle économie. Les travaux de la feuille de route pour l'économie circulaire ont confirmé qu'il est plus pertinent de définir les objectifs et non les moyens des filières REP.

avant biodégradation est très longue. Jusqu'à la fin de l'année 2018, selon la grille tarifaire de Citeo, en France, une bouteille végétale, biodégradable et compostable déclenchait un malus de 100 % par rapport à son équivalent plastique. Si ce malus a été levé en 2019, le prix de ces emballages compostables demeure largement supérieur à celui d'un emballage en plastique conventionnel. Les emballages compostables devraient, comme pour les emballages intégrant une part de matière recyclée, pouvoir bénéficier d'un tarif plus attractif que le plastique vierge. Cet amendement vise à inscrire dans la loi la compostabilité et l'absence d'écotoxicité comme critères de performance environnementale pouvant donner lieu à une prime accordée par l'éco-organisme au producteur.

parole est à M. Frédéric Marchand. Nous devons renforcer la lutte contre la pollution liée à certains déchets abandonnés au sol ou dans la nature. La modulation des contributions financières versées par les producteurs prend en considération un nombre important de critères, mais pas celui de la biodégradabilité.

On se trouve, comme nous l'avons déjà dit, dans un système où le lien qui unit les éco-organismes à ses adhérents metteurs sur le marché conduit à une confusion d'intérêt et à un mélange des genres. Pour répondre à ce problème, le projet de loi instaure un simple autocontrôle sur la gestion financière, le respect de la couverture des coûts, la mise en place d'un dispositif financier de sauvegarde, autant d'éléments qui ne sont pas suffisants. C'est bien l'ensemble du système qu'il faut repenser afin de garantir que les sommes collectées, payées par les consommateurs, serviront bien au but d'intérêt général défini par le cahier des charges des éco-organismes. Ces taxes, car il s'agit bien de cela, ne peuvent être perçues comme une fiscalité verte dont l'utilisation ne correspondrait pas aux enjeux affichés. Or la Cour des comptes n'a de cesse d'épingler ce système, qui conduit notamment les éco-organismes à des abus. Dans la droite ligne des amendements que nous avons proposés, et alors que le projet de loi permet de renforcer les modulations des éco-contributions en fonction de la performance des produits mis sur le marché, il semble nécessaire d'aller plus loin et de confier la définition de éco-modulations à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en dialogue avec le ou les éco-organismes. Nous savons que certaines associations ont proposé pour cette mission la création d'une haute autorité. Nous préférons, pour notre part, et alors que les compétences existent déjà dans la sphère publique, laisser le soin à l'Ademe de défendre ses intérêts, ce qui permet également de réinstaller cette instance dans ses missions au service de l'économie circulaire et de l'environnement.

Conformément au principe de responsabilité élargie du producteur, il est nécessaire que les producteurs assument eux-mêmes la responsabilité de la fin de vie de leurs produits et continuent de fixer ces éco-contributions, l'État conservant un regard sur ces éco-contributions

parole est à M. Frédéric Marchand. Cet amendement vise à réintroduire une disposition supprimée en commission. Le texte initial prévoyait que les modulations des éco-contributions étaient présentes dans la liste des éléments pouvant être pris en compte dans l'affichage environnemental prévu à l'article 1 du présent texte. Ne pas rendre visibles ces modulations nuirait à l'efficacité du dispositif. L'incitation financière est bien souvent faible : quand la contribution sur un vêtement est d'une fraction de centime, ou celle sur un smartphone de quelques centimes, même 100 % de bonus ou de malus n'est pas incitatif. L'effet « image » est donc important pour l'efficacité réelle de ce dispositif, c'est elle souvent qui incite les producteurs à évoluer. C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir que le producteur ou l'importateur rende accessibles au public les critères retenus pour le produit qu'il met en vente, en bonus et en malus.

Quel est l'avis du Gouvernement ? Cette information me paraît tout à fait utile pour assurer la transparence du dispositif d'éco-modulation, tout en permettant au consommateur d'être mieux informé. Nous avons eu ce débat hier : la transparence est la clé. Je suis donc tout à fait favorable

S'il est bien précisé que la prime est accordée si le produit respecte des critères de performance environnementale, la rédaction proposée en ce qui concerne la pénalité est floue, puisqu'elle serait appliquée si le produit s'éloigne de ces critères. La mention « s'en éloigne » ne constitue pas un critère d'appréciation objectif par l'éco-organisme et les autorités publiques pour contrôler l'atteinte des critères d'éco-conception définis par les textes réglementaires et les cahiers des charges des éco-organismes, comme la recyclabilité des produits, leur démontabilité ou leur réparabilité.

Sagesse.

une partie de l'éco-contribution afin de leur permettre, en fonction des territoires, de choisir une stratégie spécifique favorable pour le stockage des déchets.

Aujourd'hui, cette obligation n'existe pas. La très grande majorité des acteurs de la filière ne réincorpore donc pas ce type de fibres recyclées. Le recyclage textile n'a donc aucun effet en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur, quatrième émetteur mondial, alors que ces émissions devraient diminuer de moitié d'ici à 2030 pour rester dans un scénario de 1,5 degré et éviter l'emballement climatique. Cet amendement vise donc à prévoir au 1 janvier 2023 la réincorporation obligatoire de 10 % de fibres recyclées dans les produits mis sur le marché. Cette disposition viendra compléter les incitations financières à la réincorporation mises en place depuis 2013 par l'État, mais beaucoup trop faibles pour produire des effets.

dans les textiles pour fermer la boucle, éviter les effets rebonds et maîtriser davantage la pollution microplastique générée par les vêtements issus du recyclage de PET. Il s'agit d'un instrument indispensable dans la mesure où les incitations financières à la réincorporation mises en place depuis 2013 par l'État sont trop faibles. Je cite, par exemple, l'allégement de 50 % d'une éco-contribution, qui n'est que de 0,7 centime par vêtement et qui n'a produit aucun produit aucun effet. L'exemple de la filière plastique où les engagements volontaires des entreprises restent insuffisants, comme le reconnaît le Gouvernement, montre que les acteurs n'agiront pas suffisamment s'il n'y a pas de contrainte réglementaire. Quel est

Le projet de loi prévoit qu'une part des contributions versées par les producteurs à l'éco-organisme finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de la réparation d'un bien effectuée par un réparateur labellisé. Or les producteurs financent déjà la réparation de leurs produits. L'amendement tend, en conséquence, à ne pas mettre le financement de la réparation à la charge de l'éco-organisme, celle-ci restant directement gérée par le producteur. Quel est l'avis de la commission La commission ne peut que s'opposer à la suppression du fonds de réparation, qu'elle avait introduit dans le projet de loi à l'unanimité. Il est important de rappeler que, selon l'Ademe, le coût de réparation est le critère privilégié par 66 % des Français au moment de choisir de faire réparer ou de remplacer un produit cassé ou en panne. Seule la prise en charge d'une partie de ce coût peut donc significativement augmenter le recours à la réparation. C'est donc non seulement une mesure d'intérêt environnemental, mais aussi économique. La réparation des produits soutient en effet le pouvoir d'achat des Français.

l'amendement n° 43 rectifié. Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 541-10 du code de l'environnement introduit par l'article 8 du projet de loi, qui refonde le périmètre du principe pollueur-payeur mis en oeuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs. Ce périmètre est explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l'insertion par l'emploi ainsi qu'au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l'économie sociale et solidaire. Les associations de réemploi solidaire- Emmaüs, ressourceries, recycleries, Secours catholique, ateliers vélos, etc. -qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets- 90 % des tonnages collectés sont valorisés -et créent des milliers d'emplois pour les plus précaires : les 10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre trente et un pour le recyclage, trois pour l'incinération et un pour l'enfouissement. Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d'engagement bénévole et d'animation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu'elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d'accéder à une consommation écologique et responsable. Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales peuvent se traduire en créations d'équipements de proximité, en développement d'activité de collecte et de valorisation en réemploi et en création d'emplois par les associations mais il faut pour cela, à l'instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux. Le présent amendement vise donc à créer un fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale. l'amendement n° 133 rectifié. Nous examinons ici un amendement fondamental. Le fait qu'il soit déposé sur toutes les travées de cet hémicycle est un signe remarquable dont je me félicite. Nous avons évoqué le réemploi en début de texte, et nous avons fixé un objectif dans la loi : doubler la part de déchets réemployés d'ici à 2030.

Or leurs financements ne sont pas pérennes et sont beaucoup trop dépendants des subventions publiques, une denrée que l'on sait instable en ces périodes de disette budgétaire. Aussi, nous vous proposons que ce fonds soit financé par une ponction de 5 % des éco-contributions destinées aux éco-organismes. Ce prélèvement ne subsiste pas aux autres versements réalisés par les éco-organismes pour réemploi. Ce mécanisme s'inscrit parfaitement dans le principe de la responsabilité environnementale des entreprises et du principe pollueur-payeur. Il est on ne peut plus légitime que les entreprises financent les recycleries, les ressourceries et les associations qui donneront une nouvelle vie à leurs produits. En revanche, au regard de leur fonctionnement, il est indispensable que ce fonds soit majoritairement administré par le secteur des associations, accompagné des représentants de l'État, particulièrement des collectivités. On l'a dit et on le répète, il y a des milliers d'emplois de réinsertion à la clé, il y a des millions de tonnes de déchets à détourner des décharges et des incinérateurs. L'Ademe estime ainsi que 9,3 millions de tonnes de déchets ménagers sont réemployables, et nous en réemployons aujourd'hui quelque 900 000 tonnes, soit 2,5 % du total des déchets.

élargie du producteur permette un soutien aux réseaux de réemploi tels que ceux qui sont gérés par l'économie sociale et solidaire. S'il est une économie verte et vertueuse, anticipatrice, c'est bien celle-là ! Ces réseaux fonctionnent déjà, et ils démontrent leur capacité et leur savoir-faire. Les associations de réemploi solidaire comme Emmaüs, les ressourceries, le réseau des recycleries et maintenant les réseaux des matériauthèques ont un rôle essentiel dans la gestion des déchets. Ils ne nous ont pas attendus pour se prendre en main. Ces associations permettent par leur activité de collecte et de tri de valoriser une quantité importante d'objets, qui, sans elles, seraient venus alimenter la masse des détritus. Via cette activité, elles fournissent des milliers d'emplois, notamment pour les plus précaires. Ces associations sont des atouts indispensables pour les territoires et le développement local. Elles permettent aussi, parce qu'elles fournissent à bas coûts des biens réemployés, un accès à la consommation pour des personnes en difficulté économique, avec un impact écologique positif. Afin de développer ces activités, qui correspondent au coeur des logiques de diminution des déchets, il importe de mettre en place un financement adapté qui permettra de créer des emplois, porteurs de sens, notamment pour les personnes en insertion, ainsi qu'un maillage plus fin du territoire pour ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, vecteurs de lien social. La

Les associations de réemploi solidaire collectent, trient et donnent une grande quantité de déchets. Parmi tout cela, 90 % des tonnages collectés sont valorisés. Je ne citerai qu'un seul chiffre on ne peut plus parlant : 10 000 tonnes

plusieurs nouveaux outils destinés à financer et à soutenir des actions de réemploi, parmi lesquels, par exemple, une meilleure information des consommateurs, l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires, la refonte du fonctionnement des filières REP. REP. Je suis favorable à ce que des objectifs de réemploi et de réutilisation soient fixés aux éco-organismes et qu'ils soient sanctionnés en cas de non-atteinte de ces objectifs. L'Ademe mène aussi des actions en faveur du réemploi en s'appuyant sur le fonds déchets-économie circulaire- je pense aux appels à projets pour soutenir les initiatives des consignes locales pour réemploi. La création d'un nouveau fonds de réemploi financé par un prélèvement sur les éco-organismes tel que vous le proposez soulève certaines difficultés opérationnelles.

En outre, votre dispositif s'apparente à la création d'un prélèvement obligatoire sur les éco-organismes, qui nécessiterait un examen dans le cadre d'une loi de finances. Quoi qu'il en soit, je partage avec vous l'ambition de renforcer le réemploi et la réparation. C'est la raison pour laquelle je m'en remettrai à la sagesse du Sénat sur cette mesure, mais soyons réalistes.

notamment de réparation, un peu plus techniques. Aujourd'hui, elles n'ont pas les moyens de mettre en place des ateliers pour, par exemple, réparer l'électroménager et le proposer à la revente à des publics socialement en difficulté, qui ne peuvent pas s'acheter du neuf.

Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 541-10 du code de l'environnement

représentent une part très importante des déchets non triés actuellement par les particuliers comme par les entreprises. C'est un gisement de 8 millions de tonnes au total, soit 30 % à 40

par les éco-organismes, véritables leviers de la transition écologique, doit être consacrée à l'évolution des comportements, en incitant et facilitant le geste de tri dans le but d'obtenir un meilleur traitement de l'ensemble des biodéchets.

complexe, des oxofragmentables, des prétendus biodégradables, etc. Il y a actuellement des recherches sur des plastiques biosourcés qui sont effectivement compostables. Il faut encourager cette filière

pour développer les filières locales de recyclage des déchets et favoriser le recours aux emplois d'insertion. Il ne me paraît pas opportun de fixer un seuil plus élevé en l'absence de retour d'expérience de cette mesure. De plus, cela pourrait la fragiliser d'un point de vue juridique. Je mets aux voix

parole est à M. Frédéric Marchand. Depuis quelques mois, les mêmes images se multiplient : étouffant sous les amoncellements de plastiques, des pays d'Asie du Sud-Est ne veulent plus recevoir autant de déchets exportés depuis les pays développés. Après la Chine, la Malaisie ou encore les Philippines, l'Indonésie a récemment dit « stop La question de la traçabilité des flux de déchets est donc centrale. Lorsqu'ils sont exportés à l'étranger en vue de leur traitement, définitif ou non, les procédures prévues par les textes internationaux s'appliquent. Dans le cadre des transferts de déchets non dangereux pouvant être soumis à la responsabilité élargie des producteurs, l'accord préalable du pays d'expédition et son information préalable ne sont pas systématiquement prévus dans les textes réglementaires européens et internationaux. Il en découle un manque de connaissance des différents flux. Cet amendement a donc pour objet de créer l'obligation pour les éco-organismes de déclarer leur flux de déchets vers l'étranger et, par là même, d'améliorer leur traçabilité. Quel est l'avis de la commission

permettant un transfert de la charge des contribuables vers les producteurs. L'avis est favorable sur l'amendement n° 41 rectifié, car il est évident que les obligations de reprise par les distributeurs ne peuvent concerner que les produits authentiques. Il s'agit, bien entendu, d'exclure les contrefaçons du dispositif.

Les innovations technologiques permettent aux gestionnaires de déchets et aux collectivités territoriales compétentes d'augmenter l'efficacité du tri et d'améliorer le traitement des déchets. Par exemple, certaines colonnes de tri dotées d'une interface numérique collectent, grâce aux informations entrées par l'utilisateur dans une application mobile dédiée, des données personnelles qui peuvent être stockées, réutilisées ou transmises. Ainsi, l'analyse fournie par ces colonnes intelligentes sur les habitudes de tri et la collecte des déchets permet une anticipation et une adaptation constantes de la part des gestionnaires de déchets. Si cet objectif est louable, il ne saurait être la porte ouverte à la marchandisation du tri. En effet, les données collectées, dès lors qu'elles fournissent des informations précieuses sur les habitudes de consommation des individus, pourraient revêtir un enjeu économique non négligeable. Afin de lutter contre la captation de ces données à des fins lucratives, le présent amendement, soutenu par de nombreux collègues, notamment du groupe Union Centriste, vise à imposer le recours

du Gouvernement ? La loi Informatique et libertés met l'informatique au service de chaque citoyen, à condition, bien sûr, qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles. le principe d'interdiction de la commercialisation des données personnelles obtenues dans les colonnes de tri connectées, mais ces données peuvent fournir des informations utiles sur les habitudes des individus, notamment sur leurs gestes de tri. Leur utilisation sous forme de données agrégées et anonymes permettrait de développer la prévention et le tri de ces déchets.

Mme Nicole Duranton. Cet amendement vise à inclure dans le dispositif les nouveaux modes de transport proposés en. Ces appareils, dotés d'un mécanisme de géolocalisation, fonctionnent à l'aide de batteries contenant de multiples produits hautement inflammables, voire explosifs, tels que le lithium. Il est par conséquent indispensable d'obliger le

en France et sont une des principales sources de pollution plastique. Considérant la nécessité de lutter contre cette pollution, qui dévaste nos milieux naturels, et l'objectif fixé à l'article L. du code de l'environnement de réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers et assimilés, cet amendement a pour objet d'introduire un objectif de réduction des emballages plastiques ménagers mis sur le marché, lequel devra être précisé par décret. Cet objectif de réduction pourra être atteint par l'élimination de certains emballages, ainsi que par le développement d'emballages réemployables. Quel est

du fait de la mise sur le marché de produits générateurs de déchets : « dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé ».

qui serait contraire au principe pollueur-payeur. Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement le traitement des déchets afin d'améliorer la couverture des coûts supportés par les collectivités et de responsabiliser les producteurs de déchets.

12 000 habitants, de la Désirade, à peu près 1 500 habitants, et de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, environ 3 000 habitants. Du fait de cette double insularité, ces îles nécessitent un dispositif d'accompagnement spécifique, notamment en matière de traitement et de valorisation de leurs déchets. Cet amendement vise donc à prévoir la prise en charge financière des activités de transport des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur de ces îles vers la Guadeloupe dite « continentale » par les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe.

Je reconnais que certains éco-organismes tardent à se déployer dans les territoires d'outre-mer. C'est pour cette raison que le projet de loi prévoit que les éco-organismes doivent renforcer leur couverture des coûts supportés par les collectivités territoriales. Il dispose notamment que l'ensemble des coûts de transport sont à la charge de l'éco-organisme,

faire ? Outre l'évidente nécessité de prévention et de sensibilisation, il y a aussi des moyens de sanction modernes, qui peuvent avoir une certaine efficacité. Je n'aurais pas fait cette proposition si je n'avais pas travaillé dans le cadre de la loi sur les mobilités avec l'excellent Cerema, l'organisme d'ingénierie de l'État, qui met au point des dispositifs de vidéocontrôle basés sur le traitement d'images.

est à M. Jean-François Longeot. La récupération et l'utilisation de l'eau de pluie suscitent un intérêt croissant en France, cette ressource permettant facilement de satisfaire des besoins en eau ne requérant pas une qualité d'eau potable. Je pense, par exemple, à l'arrosage des espaces verts dans nos communes ou à la possibilité de garantir une certaine autonomie dans les périodes de sécheresse. Si un arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments autorise autorise cette utilisation des eaux de pluie à l'intérieur des établissements recevant du public, ce même texte prévoit de nombreuses exceptions ne permettant pas le développement de leur utilisation pour l'alimentation des toilettes, le lavage des sols ou encore du linge. Les utilisations sont pourtant pléthores et leur développement tient à plusieurs facteurs : des considérations environnementales, afin d'éviter de gâcher l'eau potable ; une nouvelle approche de l'aménagement, plus attentive à une gestion raisonnée des ressources, avec des matériaux limitant au maximum les pertes une plus grande reconnaissance par les collectivités, qui l'inscrivent au sein de leur agenda 21 pour satisfaire leurs propres besoins et soutenir des programmes locaux d'incitation financière à développer un tel usage. À cet égard, le présent amendement est un amendement pragmatique

parole est à M. Frédéric Marchand. Dans un contexte de raréfaction des ressources en eau douce, de moindre accessibilité, de changement climatique et de déséquilibre entre la demande et la ressource disponible, la demande de réutilisation des eaux usées traitées se fait de plus en plus pressante dans les régions en tension quantitative. Cette pratique est souvent présentée comme une solution de substitution, notamment pour l'irrigation des cultures. Elle n'est cependant pas sans conséquence sur les milieux naturels et les espaces récepteurs de ces eaux ainsi que sur la santé humaine. La directive-cadre sur l'eau de la DCE, engage les États membres de l'Union européenne à atteindre l'objectif du « bon état » des masses d'eau en 2015, avec des dérogations possibles pour 2021 et 2027. C'est un objectif ambitieux en matière de reconquête de la qualité physico-chimique et écologique des masses d'eau, de maintien et de restauration des usages liés. Cet objectif est complété par le principe de non-détérioration de l'état des masses d'eau et par celui de réduction du degré de traitement de l'eau pour la consommation humaine. Un développement rapide et sans condition de la réutilisation des eaux usées traitées pourrait nuire à l'atteinte des objectifs fixés dans la DCE et exposer l'État français à un risque de contentieux. Dans ce contexte, cet amendement vise à conditionner le développement de la réutilisation des eaux usées traitées à une compatibilité avec l'atteinte du « bon état » des masses d'eau qui figure dans la directive-cadre sur l'eau.

n° 243 rectifié. Les alinéas 6 et 7 de l'article 8, résultant de l'examen du texte par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, imposent de nouvelles contributions au titre du principe pollueur-payeur, notamment sous forme d'éco-conception, d'information du consommateur ou de contributions financières pour la mise sur le marché de matériaux et produits qui ont un impact négatif sur l'eau et les milieux aquatiques. Ces nouvelles contributions,

qui crée une nouvelle contribution financière pour les fabricants et importateurs de produits susceptibles de polluer les milieux aquatiques. Les activités économiques participent déjà au financement des mesures de préservation de la ressource en eau au travers des redevances qu'ils versent aux agences de l'eau en application du principe du pollueur-payeur. Le Gouvernement considère qu'il n'est pas souhaitable d'introduire une obligation supplémentaire qui viserait le même objectif. Quel est l'avis de la commission ? Les amendements identiques n 243 rectifié et 459 visent à supprimer un ajout inséré en commission sur l'initiative de nos collègues Didier Mandelli et Jean-Paul Prince, qui permet, en application du principe du pollueur-payeur, de faire contribuer, en nature ou financièrement, certains producteurs dont les produits ont des impacts négatifs importants sur l'eau et les milieux aquatiques. plusieurs catégories de produits contribuent de façon très importante à la pollution aquatique, tels les emballages plastiques, les produits cosmétiques et d'hygiène ou encore les médicaments. Souvent à l'origine de micropolluants difficiles à traiter par les systèmes d'épuration et d'une forte contamination des milieux aquatiques, ces produits et leurs déchets génèrent un impact négatif important sur l'environnement, lequel n'est pas pleinement assumé sur le plan opérationnel ou financier par les producteurs. En outre, cette micropollution constitue une préoccupation croissante au sein de la population. L'article 8 permet au pouvoir réglementaire d'exiger des producteurs de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ces produits sur l'eau et les milieux aquatiques. Cette contribution pourra prendre différentes formes, comme une démarche d'éco-conception, une information du consommateur ou une contribution financière à la dépollution de l'eau. Compte tenu des fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur la politique de l'eau et que déplorent de très nombreuses collectivités territoriales, un tel dispositif permettra de mettre à contribution certains pollueurs de façon juste et équitable. Par conséquent, la commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Avis favorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le code de l'environnement prévoit que la bonne gestion des déchets, dans le respect du principe de proximité, est de la responsabilité du producteur de ces déchets. Les collectivités sont uniquement responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés. Le dispositif

et facile à comprendre. Elle ne sera réalisable que lorsque l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques sera effective. Or la perspective d'une consigne a bloqué les projets de modernisation des centres de tri, retardant d'autant l'extension des consignes de tri au niveau de la collecte. De ce fait, la mise en oeuvre partielle de l'extension des consignes de tri brouille le message auprès des habitants, qui ne reçoivent pas tous les mêmes indications de collecte. Afin de leur permettre d'habituer le plus rapidement possible les habitants aux nouveaux comportements de tri, les collectivités doivent pouvoir unifier les consignes de tri dès que leurs équipements de collecte le leur permettront, sans attendre la modernisation des centres de tri. Tel est l'objet du présent amendement.

Guillaume Gontard. Par cet amendement, nous proposons d'aller dans le sens de l'article 9, qui prévoit l'obligation pour les surfaces de vente de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation de se doter d'un point de reprise des déchets d'emballage. Si nous souscrivons à cette mesure et à son objectif, à savoir faciliter le recyclage des emballages et renforcer la responsabilité des hypermarchés, nous proposons d'aller plus loin, en visant non pas les surfaces de plus de 2 500 mètres carrés, mais celles de 1 000

Cet amendement tend à élargir cette possibilité à tous les commerces de plus de 1 000 mètres carrés. Concrètement, de nombreuses grandes surfaces ont déjà mis en place des espaces de vrac pour répondre à la demande des consommateurs. Dès lors, inscrire une telle obligation dans la loi nous semble très peu contraignant pour les commerçants. Cela ne fera que donner un petit coup d'accélérateur à un mouvement déjà largement engagé.

Selon ces dispositions, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballage et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire. Cet objectif d'harmonisation nous semble important. Il suppose de la part des collectivités un effort non négligeable, puisqu'il implique notamment un renouvellement des bacs de collecte.

renforcée. En l'état, il ne s'agit nullement d'une obligation : c'est une simple faculté, fondée sur le volontariat. Par cet amendement, nous proposons donc d'accroître les responsabilités des éco-organismes en les obligeant à s'investir dans cette démarche d'harmonisation des contenants, qui répond à l'objectif d'une meilleure collecte sur l'ensemble du territoire national des déchets d'emballage et des papiers graphiques. Quel

Le Gouvernement souhaite préciser dans la loi les modalités de prise en charge des coûts supportés par les collectivités, qui assurent la collecte et le tri des déchets d'emballages ménagers papier. Le présent amendement fixe ainsi le taux de prise en charge des coûts qui devront être supportés par l'éco-organisme : 80 % pour ce qui concerne les emballages ménagers, comme c'est le cas depuis les travaux du Grenelle de l'environnement et la loi de 2009, 50 % pour ce qui concerne les déchets papier, ce qui ce qui est supérieur au taux actuel. Il s'agit là d'un enjeu essentiel, parce que c'est de ces modalités que dépend le soutien aux collectivités. La directive-cadre Déchets est en effet très claire sur ce sujet : ce sont les coûts optimisés nets de la revente des matières triées qui doivent servir de base pour le calcul des soutiens que Citeo verse aux collectivités. Ainsi, si les collectivités revendent moins de matières triées, les soutiens de Citeo doivent automatiquement augmenter pour compenser les pertes. Il s'agit d'une sorte d'assurance pour les collectivités, qu'il convient de conforter dans la loi. Aux termes de l'amendement, la couverture des coûts serait portée à 100 % pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution pour tenir compte des spécificités de ces territoires, que l'on ne peut ignorer,

suite à l'adoption en commission du renforcement de la collecte sur les emballages hors foyer, cet amendement vise à préciser que les producteurs relevant de la filière REP sur les emballages professionnels devront également contribuer à la mise en place de cette collecte sélective.

à M. Éric Gold. La collecte des produits nomades, qui sont consommés hors foyer, constitue l'un des principaux leviers pour accroître l'efficacité du service public de gestion des déchets. Aussi, nous sommes favorables à l'ajout par la commission de la mise en place d'un programme visant à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des emballages nomades. Or ce programme serait établi par les producteurs de la filière REP emballages ménagers d'ici à 2025. Nous considérons que cette date est bien trop lointaine, alors que le paquet européen Économie circulaire impose des objectifs ambitieux dès 2025.

des déchets plastiques à l'ensemble des filières REP. C'est un enjeu important.

et des emballages plastiques à usage unique en particulier soient intégrés au cahier des charges des éco-organismes. L'amendement vise en effet à préciser que cette réduction des emballages se fait notamment via le développement d'emballages réutilisables et la standardisation de ces emballages. Il s'agit ici de favoriser le succès de la consigne pour réutilisation. En effet, comme cela a déjà été dit, pour que la consigne pour réemploi soit efficace et vertueuse sur le plan environnemental, il faut limiter au maximum le transport des emballages consignés. L'Ademe a montré que le système de consigne pour réutilisation était optimal, à condition que la réutilisation s'effectue à proximité du lieu de collecte. Pour favoriser cette proximité, une solution logique est de favoriser la standardisation des emballages réutilisables. En effet, cette standardisation permet une mutualisation des emballages, mais aussi des équipements de stockage et de lavage entre les différents producteurs. C'est d'ailleurs ce que pratiquent déjà les brasseurs, notamment dans l'est de la France. L'étiquette des emballages est bien souvent suffisante pour assurer une distinction en termes de marketing. La consigne pour réutilisation est une solution d'avenir. Dès lors, il est important d'intégrer au cahier des charges des éco-organismes à la fois la notion de réutilisation des emballages et celle de la standardisation de ces emballages.

que la diminution de la mise sur le marché des emballages, en particulier des emballages plastiques à usage unique, prévue par le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés doit, pour les produits alimentaires, se faire au profit du verre. En effet, cette matière est recyclable à l'infini, moins génératrice de pollution et bien meilleure sur le plan sanitaire : les microplastiques présents dans l'eau du robinet, générés en partie par la dégradation des déchets plastiques, ne sont pas sans impact sur la santé et sur l'environnement.

La densité des corbeilles de tri dans l'espace public est largement insuffisante en France, alors qu'elles permettent à nos concitoyens de pratiquer le geste de tri à la source. Elles sont indispensables si l'on veut améliorer le taux de recyclage des produits consommés hors foyer. Et, là encore, on connaît des marges de progression. Cet amendement vise à accélérer l'installation de ces corbeilles permettant au moins de collecter séparément le plastique et le papier, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des corbeilles de propreté. En outre, il tend à permettre aux éco-organismes d'accompagner les collectivités en vue d'atteindre nos objectifs en matière de collecte et de gestion des déchets.

amendements identiques visent à accélérer l'installation des corbeilles de tri dans l'espace public. Cependant, la date du 1 janvier 2022 laisse entendre que l'accompagnement des éco-organismes va être limité dans le temps. Il est nécessaire que les collectivités puissent être accompagnées par les éco-organismes au-delà de cette date pour que le déploiement de ces nouvelles solutions de tri se fasse progressivement et efficacement. Le sous-amendement vise donc à supprimer l'échéance du 1 janvier 2022, de façon à ne pas limiter dans le temps le soutien des filières REP.

Le tri des biodéchets des ménages, notamment en zone urbaine, est très compliqué. Beaucoup d'immeubles ne sont pas en mesure d'accueillir des composteurs, faute de place ou d'aération. Beaucoup de nos concitoyens qui souhaitent recycler leurs biodéchets ne sont pas en mesure de le faire, faute de solution de compostage accessible. Cet amendement vise à renforcer le maillage des composteurs en ville en les multipliant dans les résidences, à la charge des bailleurs sociaux, dans les parcs et jardins et, surtout, dans les écoles. Il répond à une pratique vertueuse de nos concitoyens, entravée par manque de débouchés. Il répond aussi à un besoin en fumier de nombreuses communes, au premier rang desquelles la capitale. Ces dernières ont besoin d'engrais naturel pour leurs espaces verts à la suite de l'interdiction de produits phytosanitaires instaurée par l'excellente loi de mon collègue Joël Labbé. Enfin, les composts dans les écoles, phénomène déjà très répandu dans nos communes, sont utiles à la fois pour offrir des débouchés aux parents souhaitant traiter leurs biodéchets et pour l'éducation des élèves aux fondamentaux de l'économie circulaire et du jardinage. Les composts scolaires s'accompagnent souvent d'un petit potager dans les projets

présenter l'amendement n° 8 rectifié. La filière française des déchets électriques et électroniques ménagers repose depuis 2006 sur un mécanisme de transparence et d'information sincère du consommateur quant au coût de collecte, de dépollution et de recyclage des équipements. L'éco-participation est ainsi indiquée de manière visible, distincte du prix des produits, et versée à un éco-organisme qui assure un recyclage de qualité de ces déchets. Ce mécanisme a été prolongé en urgence par la loi du 24 avril 2013, déposée sur l'initiative du Sénat

Ce mécanisme, simple modalité d'affichage d'une obligation légale et reposant uniquement sur les metteurs en marché, garantit que l'éco-participation est effectivement versée aux éco-organismes en empêchant la prise de marge tout au long de la chaîne de valeur. Après treize ans de mise en oeuvre, sa remise en cause viendrait déstabiliser une filière efficace et soulèverait des enjeux financiers, alors que la filière travaille en lien direct avec les collectivités locales, lesquelles assurent 57 % des collectes dont les coûts dont les coûts sont pris en charge à 100 % par les éco-organismes. Je propose de pérenniser ce mécanisme ayant fait ses preuves afin de stabiliser une filière engagée dans un recyclage à haute valeur environnementale, à haute valeur économique, à haute valeur sociale. La parole

Dans ces conditions, la réduction du principe du pollueur-payeur à un principe du producteur-payeur est à tout le moins inéquitable si l'on considère que les décharges sauvages résultent principalement de comportements illégaux

C'est le cas de certains matériaux pour lesquels les producteurs ont, de longue date, prévu des infrastructures de collecte et de valorisation. Cet amendement vise donc à reconnaître que la résorption des décharges sauvages doit reposer sur une responsabilité collective incluant, au-delà des producteurs, l'ensemble des acteurs de la construction.

comportant de l'amiante et de savoir qui doit ventiler les coûts de remise en état de sites sur lesquels la réalité est souvent complexe avec la présence pêle-mêle de déchets inertes, non inertes, pneus, batteries, emballages ... Cet amendement vise donc

monsieur Cuypers. L'amendement n° 668 vise à revenir sur une disposition introduite en commission à un large consensus qui permet de prendre en charge les coûts associés à la résorption des dépôts sauvages issus des déchets du bâtiment

Avis défavorable.

Cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, ces derniers n'ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Le cahier des charges de la filière des emballages ménagers, par exemple, prévoit un objectif de recyclage de 75 % des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70 %. Cela s'explique notamment par le fait qu'une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n'a toujours pas de solution industrielle de recyclage- de recyclage- pots de yaourt, emballages multicouches, emballages en PVC ... La non-atteinte de cet objectif ne fait l'objet d'aucune sanction. L'éco-organisme n'a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances.

Parlement afin de mieux caractériser le dépôt sauvage et de hiérarchiser les besoins en résorption et en dépollution des sols et leurs coûts associés. Ce dispositif permettrait de proratiser les contributions financières de chaque branche à hauteur des dommages environnementaux qui lui sont imputables, car les déchets du bâtiment représentent une faible part des dépôts sauvages par rapport à l'abandon d'autres déchets tels les pneus ou les batteries, par exemple.

L'établissement de ce rapport passerait forcément par une sollicitation des collectivités locales pour obtenir des informations et des données sur leur action, alors même qu'elles travaillent d'arrache-pied pour résorber les dépôts illégaux. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

et solidaire. En vertu de l'article 40 de la Constitution, les parlementaires ne peuvent procéder eux-mêmes à la création d'une Autorité administrative indépendante ni accroître les missions d'une AAI existante. Cet amendement vise à solliciter du Gouvernement la remise d'un rapport évaluant l'opportunité d'améliorer la régulation des filières REP détaillant les moyens d'y parvenir. Plusieurs situations récentes ont montré les limites de l'encadrement actuel des filières REP. C'est le cas notamment dans la filière du recyclage des panneaux photovoltaïques, dans la filière des déchets dangereux des ménages ou encore dans celle des meubles usagés. C'est véritablement très grave. La création d'une instance indépendante pourrait permettre d'équilibrer le rapport de force au sein des filières REP, très souvent à l'avantage des metteurs en marché, et de soutenir les services du ministère de l'environnement dans leur rôle d'arbitre des filières REP.